divers et variés, d'avoir accès à l'information par des abonnements à des, notamment, nous avons besoin de protection, de droits effectifs ayant une portée réelle, et non partielle. Le droit à l'oubli en est un. Nous devons Nous devons avoir le droit, indépendamment de notre âge au moment de la collecte des données, d'effacer les empreintes que nous laissons sur la toile, dès lors que cette volonté ne porte pas atteinte à d'autres enjeux rappelés précédemment et qui figurent, d'ailleurs, à l'article 40 de la loi Informatique et libertés. En définitive, ce qui me paraît étrange, c'est que les modalités d'encadrement de ce droit sont déjà inscrites dans la loi. En faire usage ne risque donc pas de limiter d'autres droits et d'autres libertés fondamentales. En revanche, ne pas lui conférer une pleine portée est regrettable, car cela revient à affaiblir la protection des données et, par conséquent, le respect de la vie privée. Quel est l'avis de la commission ?

En 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé, dans son arrêt qu'un célèbre moteur de recherche entrait dans le champ de la directive de 1995 sur le traitement des données personnelles. Dès lors qu'ils proposent des contenus publicitaires à partir de l'indexation des sites, les moteurs de recherche réalisent un traitement de données à caractère personnel. Il s'ensuit que la CJUE a reconnu la possibilité pour tout internaute d'obtenir qu'un lien n'apparaisse plus quand son patronyme, et uniquement son patronyme, est saisi sur le moteur de recherche. C'est le droit au déréférencement. Ce droit est naturellement à mettre en balance avec d'autres impératifs, tels que le droit à l'information du public. Pour autant, une question n'a pas été arbitrée : quelle en est la portée territoriale ? Autrement dit, lorsqu'un moteur de recherche est tenu de déréférencer, doit-il le faire uniquement dans la zone géographique couverte par le texte réglementaire- dans notre cas, l'Union européenne -ou doit-il le faire à l'échelle mondiale, partant du postulat que, Internet étant un monde ouvert, indifférent aux frontières, l'information demeurerait accessible ? Prenons un exemple concret. Si je demande à un moteur de recherche de déréférencer un lien

en « .com ». Le droit au déréférencement est par conséquent aujourd'hui limité territorialement. D'ailleurs, la CNIL souhaite étendre sa portée. Son raisonnement est que les moteurs de recherche, ayant souvent choisi d'avoir un traitement mondial, doivent, dès lors que le droit au référencement est appliqué, le rendre

le droit au déréférencement n'est que parcellaire ! Certes, des questions préjudicielles sur ce point fondamental ont été soumises par le Conseil d'État à la Cour de justice de l'Union européenne. Toutefois, à défaut d'anticiper les décisions de la CJUE en intégrant d'ores et déjà une disposition dans notre ordre juridique interne, nous aimerions au moins connaître la position du Gouvernement sur la question. Celui-ci

est l'avis de la commission ? Comme le droit à l'oubli, le droit au déréférencement sur les moteurs de recherche est l'un des nouveaux droits garantis par le règlement général sur la protection des données. Il a vocation à s'appliquer directement, dans ce cadre, à compter du 25 mai Le problème des extensions des noms de domaine sur lequel il s'exerce ne peut être tranché par un simple ajout dans la loi nationale. En effet, les autorités de contrôle européennes sont en train de se forger une doctrine, exprimée au sein du groupe qui les rassemble,

Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel. Dès lors, seule la faculté de s'opposer à l'installation de ces compteurs

et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce règlement consacre le principe selon lequel le consentement des personnes au traitement de leurs données personnelles doit être donné par un acte positif clair, par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel la concernant. Un refus de la part de certains utilisateurs que leurs données personnelles soient collectées par les dispositifs de comptage et l'impossibilité, partant, d'installer ces dispositifs chez ces utilisateurs n'entraînera pas une violation de la directive européenne du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors que son annexe I n'impose qu'une couverture du territoire national à hauteur de 80 %.

garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement souhaite la suppression de la condition d'agrément qu'a introduite la commission pour les associations souhaitant exercer une action de groupe. Une telle condition n'est pas prévue à l'article 80 du règlement, qui vise les organismes, organisations ou associations à but non lucratif ayant été valablement constitués conformément au droit d'un État membre.

l'agrément préalable, entraverait la possibilité d'exercer ces actions. Je rappelle que la loi de 2016 a déjà prévu un certain nombre de garde-fous. En effet, pour pouvoir exercer une action de groupe, une association doit être régulièrement déclarée depuis cinq ans au moins et justifier d'un objet statutaire concernant la protection de la vie privée et la protection des des données à caractère personnel. Les associations de défense peuvent également exercer une telle action lorsque le traitement de données à caractère personnel affecte des consommateurs. L'agrément prévu pour ces associations par l'article L. 811-1 du code de la consommation est facultatif. Il y aurait donc, si nous n'avions pas déposé notre amendement, une distorsion entre ces deux types d'association. J'ajoute enfin que le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur la disposition introduite par votre commission, qui a reporté au au 25 mai 2020 l'entrée en vigueur de l'action de groupe. Au total, il nous semble que la crainte d'un déferlement d'actions en réparation apparaît excessive et que le texte est parvenu à un juste équilibre. Pour l'ensemble de ces raisons, je vous demande donc de bien vouloir adopter cet amendement de suppression,

de plaideurs virulents ayant des visées politiciennes ... Nous ne les avons pas vus à l'oeuvre jusqu'à présent ! Il nous semble donc que toutes ces préventions sont superflues et infondées. C'est pour cette raison que nous demandons la suppression des alinéas 7 à 10 de

La commission a accepté le principe de l'extension de l'action de groupe en matière de données personnelles à la réparation des dommages matériels et moraux, ainsi que l'a proposé l'Assemblée nationale. Cette extension donnera effectivement du sens à l'action de groupe en matière de données personnelles. Une action de groupe limitée à la cessation d'un manquement n'a que peu de sens, comme le Sénat l'avait relevé lors de l'examen de la loi de modernisation de la justice du XXI siècle. Telle est la véritable raison pour laquelle il n'y a eu aucune action de groupe en la matière depuis 2016. Dès lors que l'objet de l'action de groupe est étendu à la réparation des dommages, de telles actions risquent au contraire de se multiplier. C'est une grande crainte de nos collectivités territoriales.

De plus, je ne pense pas que ce soit une demande exorbitante, dans la mesure où c'est déjà le cas en matière de consommation, d'environnement, de santé. Cela permettrait aussi d'unifier le régime de l'action de groupe. La commission émet donc un avis défavorable

de rembourser à l'association ou à l'organisation mandatée les frais qu'elle a engagés. La commission ne peut y être favorable, pour plusieurs raisons : d'une part, la CNIL n'est pas une juridiction, susceptible de condamner aux dépens

Je tiens à remercier les députés et les sénateurs qui se sont mobilisés sur ce sujet, en particulier Éric Bothorel, à l'Assemblée nationale, et, au Sénat, M. Raynal et toute la commission des lois. Le Gouvernement a entendu les craintes, et nous avons travaillé longuement pour parvenir à une proposition équilibrée. Nous avons examiné avec attention les propositions qui ont été avancées en ce sens, notamment celles qui résultent de l'article 17 adopté par la commission. Cependant, sa rédaction ne nous semble ni satisfaisante ni opérationnelle, pour plusieurs raisons, mais, comme nous partageons cette ambition, nous allons vous proposer- c'est tout l'objet de cet amendement -une solution que nous trouvons acceptable et équilibrée. En premier lieu, le dispositif prévu apparaît trop éloigné, dans certains de ses énoncés, du vocabulaire même et de la logique du règlement général de la protection des données. Prenons pour exemple les notions d'utilisateur final, de nullité du contrat ou de tiers. La rédaction de l'article 17 implique en effet des acteurs tiers qui n'ont aucune obligation directe en matière de données personnelles vis-à-vis des utilisateurs finaux, sauf s'il s'agit, d'une part, de responsables ou coresponsables de traitements, et, d'autre part, de personnes concernées, au sens du RGPD, ce qui n'est pas le cas. Il serait problématique et disproportionné d'inclure l'ensemble des fabricants de terminaux dans le champ du RGPD.

le droit de la concurrence. Ce sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement, qui comprend et partage les préoccupations du Parlement, souhaite amender l'article 17 , afin de rester en cohérence à la fois avec le RGPD et avec les normes de l'Union, de façon à pouvoir conserver le dispositif dans la loi et à assurer son opposabilité aux tiers. À cette fin, l'amendement vise d'abord à mieux préciser les traitements dont il s'agit, ceux qui sont donc fondés sur le consentement, et ensuite à reprendre la logique de responsabilisation du responsable de traitement, telle qu'elle est établie

d'introduire un nouvel article dans le code de commerce prohibant « l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché des services de communication au public en ligne ayant pour objet ou pour effet de subordonner

mettant en jeu des interactions sur deux marchés distincts au sens du droit de la concurrence : le marché des services en ligne, d'une part, et celui des terminaux, d'autre part. Il vise à prohiber les abus de position dominante ayant pour effet d'imposer au consommateur d'acheter des matériels informatiques dotés

en particulier dans le cas des services accessibles des terminaux mobiles. Toutefois, nous estimons que la mesure proposée est inadéquate pour atteindre cet objectif. Oh ! Le présent amendement est malheureusement sans rapport avec l'objet du projet de loi. La modification envisagée vise à prohiber une pratique anticoncurrentielle. Elle est donc encadrée par le droit de la concurrence ; elle ne vise pas à garantir le consentement du consommateur au sens même du règlement. En outre, si nous allons au fond de l'analyse, la proposition que vous formulez pourrait laisser entendre que d'autres pratiques mises en oeuvre par ces mêmes acteurs de l'économie numérique,

En effet, alors que le consentement de l'utilisateur doit être libre et que le législateur doit s'assurer que cette liberté est totale et résulte d'un choix effectif, ce choix est en réalité limité à l'acceptation ou au refus des traitements de données ou, en l'espèce, des moteurs de recherche proposés.

La plupart de ces appareils commercialisés en France et en Europe sont en effet équipés d'un système d'exploitation mobile qui impose le même moteur de recherche- Google pour ne pas le citer. C'est une obligation faite à l'ensemble des utilisateurs. Pourtant, certains moteurs de recherche proposent des fonctionnalités équivalentes tout en offrant une meilleure protection des données. Ils s'engagent d'ailleurs sur ce sujet. C'est par exemple le cas des moteurs de recherche alternatifs,

par une entreprise d'une position dominante sur le marché des services de communication publics en ligne lorsque cette position dominante subordonne la vente d'un équipement à l'achat d'un service. En cela, monsieur le secrétaire d'État, nous sommes tellement proches des positions du ministre Bruno Le Maire ! La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

est purement scandaleuse : quelque 50 millions d'utilisateurs de Facebook se sont vu hacker leurs données par une entreprise de gestion des data, qui les a revendues

est à M. Jérôme Durain. Le paragraphe IV de l'article 18 supprime à l'article 42 de la loi du 6 janvier 1978 le caractère indirect de l'exercice des droits d'accès, de rectification et d'effacement pour les traitements de police judiciaire. Le caractère indirect est maintenu pour les seuls traitements mis en oeuvre par les administrations publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public qui ont pour mission de recouvrer des impositions. Le maintien de l'accès indirect pour cette catégorie de traitements n'est pas justifié. Il convient de prévoir que la personne intéressée peut directement exercer ses droits d'accès direct auprès du responsable du traitement de l'administration fiscale, sans passer par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Tel est l'objet du présent amendement, qui tend à abroger l'article 42 de la loi de 1978. Quel est l'avis de la commission ?

cette autorisation préalable n'est nullement exigée par l'article 28 de la directive, qui prévoit des garanties suffisantes pour la protection des droits et des libertés des personnes concernées Le projet de loi exige ainsi la réalisation d'une analyse d'impact dès lors que le traitement est susceptible de créer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment chaque fois qu'il porte sur des données sensibles.

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a choisi de maintenir un niveau élevé de protection des données personnelles en matière pénale, en conservant le régime d'autorisation préalable qui existe actuellement. La commission considère que la simple possibilité de réaliser une analyse d'impact laissée à l'appréciation des personnes morales n'est pas une garantie suffisante s'agissant de fichiers en matière pénale. Je rappelle que le considérant 15 de la directive affirme que « le rapprochement des législations des États membres ne devrait pas conduire à un affaiblissement de la protection des données à caractère personnel qu'elles offrent » et qu'il convient que « les États membres ne soient pas empêchés de prévoir des garanties plus étendues que celles établies dans la présente directive. l'invitation du Conseil d'État, l'article 19 du projet de loi maintient désormais une autorisation préalable pour les seuls fichiers mis en oeuvre pour le compte de l'État. Il convient également de maintenir ce régime pour les fichiers mis en oeuvre par les autres personnes morales, qui peuvent être tout aussi dangereux pour les droits et libertés des personnes. La commission des lois a estimé que, en matière pénale, tout fichier entrant dans le champ d'application de la directive doit être autorisé préalablement : le droit actuel doit être maintenu et non affaibli

devant être réalisée préalablement au traitement par le responsable. En effet, le contenu de l'analyse d'impact exigé par l'article 27 de la directive diffère de celui qui est prévu par le règlement. Ainsi, la directive n'impose pas une description systématique des finalités du traitement, ni une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard de ces finalités.

Je reste inquiète quant à l'absence de définition législative du contenu de l'analyse d'impact, mais je comprends la volonté du Gouvernement de la préciser par décret plutôt que par renvoi au règlement européen.

Mme Esther Benbassa. Nous nous réjouissons que ce projet de loi ait été amélioré lors de son examen par la commission des lois, notamment avec l'ajout d'un volet propre aux collectivités territoriales. En effet, initialement absentes du projet de loi, ces dernières sont largement concernées par le traitement des données personnelles, puisqu'elles gèrent en leur sein de nombreux fichiers donnant lieu à de nombreuses obligations lourdement sanctionnées en cas de non-respect. C'est pourquoi nous proposons, avec cet amendement, que soient clarifiées les modalités de saisine de la CNIL. L'alinéa 15 de l'article 19 permet actuellement aux responsables de traitement ou sous-traitants de consulter la CNIL préalablement au traitement de certaines données à caractère personnel. Nous souhaitons, et relayons en cela une attente de l'Assemblée des départements de France, que cette consultation de la CNIL soit assortie d'un avis de cette même commission, afin que les collectivités territoriales, notamment, soient épaulées et sécurisées dans leurs activités de traitement le traitement de données personnelles. Dans

Le nouvel article 70-8 inséré dans la loi du 6 janvier 1978 par l'article 19 du présent projet de loi prévoit que les données à caractère personnel figurant dans les traitements en matière pénale mis en oeuvre par les autorités compétentes devront, « dans la mesure du possible », distinguer celles qui sont fondées sur des faits de celles qui reposent sur des appréciations personnelles. Plus qu'un principe général, l'exactitude des données est un principe fondateur du droit de la protection des données personnelles. Le 4° de l'article 6 de la loi Informatique et libertés, qui définit les conditions de licéité d'un traitement de données à caractère personnel, précise qu'un traitement ne peut porter que sur des données à caractère personnel « exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour ». Il impose en outre que des mesures appropriées soient prises pour que les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées soient effacées ou rectifiées. Il est impératif en matière pénale, pour les traitements mis en oeuvre par la police et les autorités judiciaires, de distinguer les données à caractère personnel fondées sur des faits de celles qui reposent sur une appréciation subjective. Quel est l'avis de la commission ? Je partage pleinement l'objectif des auteurs de cet amendement, à savoir garantir le principe d'exactitude des données et différencier les données fondées sur des faits de celles qui sont fondées sur des appréciations. Néanmoins, la suppression des mots : « dans la mesure du possible » me semble, en l'espèce, difficile à appliquer en pratique.

du fait de la multiplication des renvois au règlement, au code pénal et à la loi du 27 mai 2008. En outre, les précisions qui sont apportées sur le profilage discriminatoire apparaissent insuffisantes, car elles ne renvoient pas à la totalité des dispositions pénales

? Il s'agit encore une fois du problème du profilage. La commission des lois, dans un souci d'harmonisation entre le droit national et le droit européen, a choisi de renvoyer à la définition du profilage donné par le règlement général sur la protection des données. Ce règlement définit le profilage comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique de cette personne physique ». La définition proposée par le Gouvernement est la suivante : « Un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne personne ». La rédaction votée par la commission est plus complète, donc plus protectrice des libertés individuelles. Surtout, le Gouvernement n'a pas transposé un point essentiel de la directive,

sceaux. Le présent amendement vise à rétablir l'obligation de moyens imposée par la directive aux autorités compétentes en matière de vérification des données avant leur transmission ou mise à disposition. La directive impose en effet aux autorités compétentes de vérifier, dans la mesure du possible, la qualité des données. Leur imposer une obligation de résultat, telle qu'elle a été adoptée en commission des lois, m'apparaît disproportionné, car cela impliquerait que la transmission de bonne foi d'une donnée qui ne serait plus à jour, y compris dans les cas où l'autorité compétente ne pouvait pas le savoir,

pourrait engager la responsabilité du gestionnaire de casier, si cette fiche n'est pas à jour des condamnations, alors même qu'un délai de quelques semaines existe entre leur prononcé par une juridiction et leur inscription au casier. Le rétablissement de l'obligation de moyens prévu par la directive paraît d'autant plus justifié que le projet de loi fixe des garanties pour s'assurer de la fiabilité des délais. En particulier, dès que l'autorité compétente prend connaissance de l'inexactitude d'une donnée transmise, elle doit en aviser le destinataire. Quel est l'avis de la commission ? l'avis de la commission ? Cet amendement tend à revenir sur l'obligation, pour les services, de vérifier la qualité des informations avant leur transmission à des tiers. Contrairement à ce qui est avancé dans l'objet de l'amendement, il ne s'agit pas ici de sanctionner les erreurs de bonne foi. Néanmoins, il est évident qu'au moins avant transfert des données, leur qualité et, surtout, leur légalité soient examinées, et cela de façon très sérieuse. Considérer une telle obligation disproportionnée semble suggérer que

résultat, imposée par la directive aux responsables de traitement dans la distinction des données en fonction des différentes catégories de personnes concernées. Imposer au responsable du traitement de tout mettre en oeuvre pour distinguer les données selon que la personne concernée est mise en cause dans une procédure pénale, coupable, victime ou tiers à une infraction pénale, constitue une stricte transposition de la directive une garantie suffisante pour les personnes. Maintenir l'obligation de résultat adoptée par la commission des lois paraît, je crois, excessif. Une telle obligation reviendrait par exemple à à pouvoir reprocher un manquement à un responsable de traitement qui n'aurait pas été immédiatement informé de ce que la personne initialement suspectée d'être l'auteur d'une infraction a été ensuite mise hors de cause et est donc devenue un tiers à l'infraction pénale.

mis en cause. Pourtant, les durées de conservation et même les droits diffèrent en fonction de la qualité de ces personnes, selon qu'elles sont victimes ou mises en cause. Il semble donc évident de prévoir que ces fichiers doivent rigoureusement distinguer la qualité de ces personnes. En conséquence,

ont à traiter, dans leurs différents services, de nombreux fichiers de données pouvant regrouper toutes sortes d'informations, y compris les plus sensibles sur nos concitoyens. De nombreuses étapes sécuritaires doivent déjà être respectées, et les fonctionnaires et agents de ces collectivités s'interrogent sur les nouvelles obligations à respecter, qui s'ajoutent à celles déjà existantes. C'est pourquoi, en portant une autre recommandation de l'Assemblée générale des départements, nous vous proposons de clarifier cette question de la sécurité des données à leur échelle. Les dispositions de cet amendement permettent ainsi au responsable de traitement de ne pas occulter les différentes obligations qui lui incombent déjà. À titre d'exemple, comme l'énonce l'objet de notre amendement, le secteur public doit aujourd'hui respecter le référentiel général de sécurité pour les hébergeurs de données de santé, ainsi que les exigences de l'ASIP Santé, entre autres. Qu'en sera-t-il avec les nouvelles règles qui incomberont aux services concernés ? Aussi apparaît-il nécessaire de préciser que le respect des nouvelles règles adaptées à notre droit européen se fasse sans préjudice des obligations nationales existantes liées à la sécurité des traitements. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Maryse Carrère. Comme je le soulignais hier lors de la discussion générale et pendant l'examen de l'article 8, le RGPD introduit une nouvelle répartition des compétences entre autorités de contrôles européennes potentiellement déstabilisatrices. Nous craignons notamment que la gestion des données personnelles ne soit traitée dans des États membres ayant choisi, dans les marges de manoeuvre laissées par le RGPD, les solutions les moins protectrices pour les données personnelles. Sans une coopération efficace entre autorités de contrôles, cela pourrait donner lieu à un affaiblissement de la protection effective des données personnelles de nos concitoyens, si la gestion de leurs données aujourd'hui traitées en France venait à être délocalisée. C'est pourquoi nous proposons de renforcer le droit d'information des personnes concernées, en prévoyant qu'elles pourront être informées de l'identité des sous-traitants et de leurs coordonnées, ainsi que des stipulations du contrat de sous-traitance relatives à la protection des données.

Il ne paraît dès lors pas cohérent de fixer un régime différent pour ces deux instruments pourtant identiques, en exigeant des seules autorités compétentes dans le champ de la directive, et non des entreprises, la transmission de ces coordonnées. Par conséquent, le

amendement vise à supprimer le délai d'un mois imposé au responsable de traitement pour rectifier ou effacer des données à caractère personnel qui a été ajouté par la commission des lois. En effet, la directive ne fixe pas de délai butoir. En outre, une échéance à un mois risque de poser d'importantes difficultés pratiques, dès lors que son point de départ n'est nullement précisé et qu'un mois paraît bien trop court pour permettre au responsable de traitement d'obtenir des informations nécessaires au traitement de la demande, puis de procéder aux rectifications ou aux effacements nécessaires. Enfin, tant le délai imparti au responsable de traitement pour répondre aux demandes de rectification ou d'effacement adressées sur le fondement du décret d'application de la loi de 1978, qui est imparti au ministère public ou à une juridiction pour statuer sur toute demande qui leur est adressée, sont de deux mois. Le délai de réponse du responsable de traitement aux demandes formées sur le fondement de la directive pourra être fixé dans le décret. Quel est l'avis de la commission ?

En l'état actuel du droit, une distinction est opérée selon que ces authentifications biométriques sont stockées dans l'appareil ou depuis des serveurs distants. Dans le premier cas, la CNIL considère que le stockage de donnée biométrique est couvert par l'exemption domestique ; dans le second cas, en revanche, la CNIL exigeait une demande d'autorisation préalable du fournisseur de l'application ou de l'appareil, en raison des risques particuliers liés à un stockage externe. Bien souvent, le consommateur ignore si les technologies d'authentification biométrique auxquelles il recourt sont stockées sur l'appareil ou sur un serveur distant. Bien souvent, les informations disponibles en ligne sur les sites des constructeurs ne sont pas suffisamment précises pour comprendre les modalités de stockage de ces données sensibles. Cet amendement vise donc à ouvrir un droit de rectification aux personnes constatant le stockage de leurs données biométriques sur un serveur distant. Quel est l'avis de la commission ? Cet amendement tend à instaurer, en matière pénale, pour les traitements concernés par la directive, un droit à l'effacement des données biométriques légalement stockées sur des serveurs distants. De surcroît, le responsable de traitement devrait pouvoir les effacer dans un délai de Je comprends très bien l'intention qui sous-tend cet amendement, mais je ne suis pas sûre que ce délai soit réaliste. Et sur quel principe fonder ce droit à l'effacement de données légalement collectées et traitées ? En tout état de cause, il ne peut y avoir un droit généralisé à l'effacement des données biométriques légalement stockées en matière pénale.

: La parole est à Mme la garde des sceaux. Cet amendement a pour objet de revenir sur la modification, adoptée par la commission des lois, exigeant que, dans le cadre du droit à l'information, le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité de former un recours juridictionnel.

Les garanties offertes à la personne concernée en cas de restriction de son droit à l'information ne sont pas pour autant réduites, puisqu'elle pourra exercer ses droits par l'intermédiaire de la CNIL, puis, en cas de refus de sa demande par cet intermédiaire, former le cas échéant un recours juridictionnel.

qui ont été opportunément écartées de la discussion jusqu'ici. Permettez-moi de vous rappeler que l'article 1 de la directive 2016/680 définit son champ d'application comme couvrant tout « traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales Il précise explicitement que font partie de ces traitements ceux qui concernent « la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ». Seules les activités relatives à la sécurité nationale ne relèvent pas du champ d'application de la directive. C'est cet argument qui nous sera opposé : la lutte contre le terrorisme, premier objectif de la loi sur le renseignement, relèverait de la sécurité nationale et ne serait donc pas concernée par les mesures protectrices instituées Cet argument, mes chers collègues, est quelque peu fallacieux. Nous le savons, l'Union européenne et ses États membres ont systématiquement considéré que la lutte contre le terrorisme entrait dans le champ d'application du droit de l'Union, prenant de nombreux actes européens à son sujet. La dernière directive 2017/541 « relative à la lutte contre le terrorisme » en est un exemple manifeste. Nous proposons en conséquence de mettre en conformité le code de la sécurité intérieure avec la directive 2016/680 et de préciser que, lorsque la mise en oeuvre d'une technique de recueil de renseignement prend fin, le service qui l'a réalisée informe promptement la personne concernée de la nature et de la durée de la technique, du type et du volume de renseignements recueillis et de la finalité

l'avis de la commission ? Cet amendement vise à étendre le pouvoir de contrôle de la CNCTR sur les données communiquées par les services étrangers. Or ce contrôle a été explicitement restreint par la loi de 2015 pour des raisons évidentes de coopération entre les États. Si nous souhaitons que nos partenaires nous transmettent des informations, il n'est pas raisonnable de multiplier les personnes ayant accès à celles-ci. Aussi, la

Le travail de renseignement ne peut s'inscrire, ce me semble, que dans un impératif de confidentialité. À l'inverse, le dispositif que vous envisagez serait de nature à vider les techniques de renseignement de leur substance, et donc à anéantir le travail des services de renseignement. Pour ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.

est à Mme Esther Benbassa. Mes chers collègues, dans le même sens que l'amendement précédemment défendu, le présent amendement vise à mettre le code de la sécurité intérieure en conformité avec la directive, laquelle est plus protectrice des libertés fondamentales de nos concitoyens. En matière de contrôle, la directive contient deux exigences. D'une part, il convient que, dans chaque État membre, une autorité indépendante contrôle l'application des dispositions adoptées en application de [cette] directive et de ses mesures d'exécution et veille au respect de celles-ci ». En France, en matière de renseignement, cette autorité de contrôle est la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. D'autre part, que « chaque État membre prévoit, par la loi, que chaque autorité de contrôle dispose de pouvoirs d'enquête effectifs. Ces pouvoirs comprennent au moins celui d'obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant l'accès à toutes les données à caractère personnel qui sont traitées. » Toutefois, en l'état actuel de notre droit, la CNCTR ne peut pas avoir accès aux renseignements collectés, exploités, échangés ou conservés par les services français, dès lors que ces renseignements ont initialement été « communiqués par des services étrangers ou par des organismes internationaux ». Bien sûr, cette disposition empêche entièrement la CNCTR de vérifier que les données personnelles collectées et exploitées par les services le sont de façon licite. Elle entre en totale contradiction avec les exigences de la directive et doit donc être corrigée. Tel est l'objet de cet amendement. Quel est l'avis de la commission ?

Dans la lignée des amendements précédents, nous souhaitons, une nouvelle fois, garantir les droits de nos concitoyens, en l'espèce le droit à un recours effectif. L'article 54 de la directive 2016/680 exige, sans aucune exception possible, que les États membres offrent aux particuliers une voie de recours juridictionnel pour contester la licéité d'un traitement portant sur leurs données personnelles. En contradiction avec cette disposition, l'article L. L. 854-9 du code de la sécurité intérieure prévoit que, en matière de surveillance internationale, les particuliers ne peuvent pas agir en justice pour contester la licéité d'une mesure

est l'avis de la commission ? La directive ne concerne que les fichiers de données personnelles et non la mise en oeuvre de techniques de recueil de renseignements.

avec le droit européen, cet amendement tend à offrir des garanties en matière de transfert des renseignements. En effet, le code de la sécurité intérieure n'impose aujourd'hui

à la directive, qui impose des normes en matière de transfert de renseignements hors Union européenne, mais aussi à notre propre droit : ce que les échanges de données avec des autorités françaises, européennes ou hors Union européenne obéissent à l'un des intérêts fondamentaux de la Nation, et que la CNCTR soit en mesure d'en assurer le contrôle. Nous proposons, en conséquence, de modifier le code de la sécurité intérieure en ce sens. Quel la commission ? La directive ne s'applique pas aux fichiers de renseignement à finalité mixte des services spécialisés de renseignement. Choisir d'appliquer de telles restrictions aux échanges entre services de renseignement ne pourrait qu'affaiblir la coopération entre

qui s'élèverait, au total, à 170 millions d'euros. Cette dotation serait compensée par la hausse de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques. Le Gouvernement vous demande de revenir sur la création de ce fonds, et ce pour plusieurs raisons.

peut susciter des interrogations : quelle serait l'équité d'un versement de cette nature ? Ensuite, cette dotation entrerait dans le périmètre des concours financiers, tel qu'il est défini à l'article 16 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, lequel comprend les prélèvements sur recettes. Or ce même article a fixé un plafond annuel de l'ensemble des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Ce montant est globalement stable jusqu'en 2022.

afin de respecter le plafond prévu par la loi de programmation. Les concours susceptibles d'être réduits à ce titre pourraient être, par exemple, les dotations de soutien à l'investissement local, la dotation globale de fonctionnement,

Pourtant, elle ne s'appliquerait qu'à partir de l'exercice 2019. Or- nous n'avons cessé de le dire depuis hier -ce règlement doit entrer en vigueur au 25 mai 2018. Depuis 2004, les collectivités territoriales sont, en tant que responsables de traitement, déjà soumises à des obligations en matière de protection des données. Nous l'avons rappelé hier, et plusieurs d'entre vous l'ont souligné.

dont la Commission européenne a estimé, dans son étude d'impact, qu'elle représente un coût unitaire de 200 euros : ce n'est pas négligeable. Je songe également à la suppression du régime d'autorisation par arrêté des traitements destinés

J'ai déjà évoqué le regard tout à fait favorable que le Gouvernement porte sur plusieurs mesures proposées par la commission des lois pour accompagner les collectivités locales.

de 1978 s'applique dans les meilleures conditions possible partout, dans tous les territoires. Il n'en demeure pas moins que le Gouvernement n'est pas favorable à l'établissement de la dotation ici proposée. Ce dispositif conduirait à réduire les dépenses nécessaires à d'autres politiques publiques menées par les collectivités territoriales.

l'objet de votre amendement : « Ainsi, cette nouvelle dotation d'un montant financier élevé, estimé à 170 millions d'euros, n'apporte aucune garantie quant à une prise en charge effective des besoins des collectivités.

disons honnêtement les choses : il n'y a pas de transfert de charges, il y a une obligation. Est-il raisonnable et responsable que le Sénat ne défende sur ce point que les collectivités ? Il faudrait aussi abonder aux dépenses des entreprises et des autres acteurs concernés. Allons au bout de notre logique, soyons honnêtes ! Je mets aux

Le manque de compétences informatiques au sein des collectivités territoriales, notamment des plus petites d'entre elles, rend cette transition d'autant plus difficile qu'elle les place dans une situation peu favorable pour évaluer le coût réel des services proposés pour le traitement de données personnelles. Dans certains cas, les relations avec les éditeurs de logiciels sont également la source de difficultés, qui rejoignent le problème plus général de détermination du prix d'un marché public.

À titre liminaire, il convient de relever que cet article modifie l'économie des dispositifs de mutualisation. On peut s'interroger sur le lien qu'il présente avec le texte en discussion, qui est relatif à la protection des données. Sur le fond, l'article 19 opère des modifications qui posent des difficultés au regard des objectifs d'intégration communautaire. Premièrement, ce nouvel article modifie la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5111-1 du CGCT, afin de permettre la conclusion de conventions de prestations de services entre, d'une part, des communes et des syndicats intercommunaux, et, d'autre part, une commune et un syndicat mixte. L'article 19 concourt ainsi au maintien d'un syndicat inclus dans un EPCI à fiscalité propre, au lieu de privilégier des transferts de compétences du syndicat au bénéfice de l'EPCI à fiscalité propre dont sont membres les communes contractantes. Dès lors, par cet article, la loi encouragerait de telles formules, alors que, au travers des schémas départementaux de coopération intercommunale, de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010 et de la loi Nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, le législateur a souhaité à l'inverse renforcer l'intégration communautaire et la diminution du nombre de syndicats.

Ces assouplissements envisagés sont de nature à aller à l'encontre de la logique de l'intégration communautaire, les transferts de compétences constituant le mode de relation privilégié entre les communes et les intercommunalités, de nature à sécuriser les actes et interventions.

en permettant la création d'un syndicat mixte ouvert associant des communes et les EPCI dont ils sont membres. Je souhaiterais enfin rappeler qu'il existe aujourd'hui de très nombreux dispositifs de mutualisation, qui sont d'ailleurs rappelés par une circulaire du 30 novembre 2015 de la Ainsi, le droit des mutualisations est un sujet vraiment complexe, qui mérite sans doute que l'on s'y attarde beaucoup plus longuement qu'au travers d'un amendement sur un projet de loi traitant de toute autre chose. Je sais que mon collègue ministre d'État, ministre de l'intérieur souhaite faire avancer ce dossier dans le cadre de la prochaine réunion de la conférence nationale des territoires, qui est prévue dans les mois prochains. Il me semble préférable de traiter ce sujet dans ce cadre général plutôt qu'à l'occasion de l'examen de ce projet de loi.

les utiliser, même si elles sont très peu nombreuses à le faire en France. Certaines communes sont proches de syndicats mixtes déjà existants, d'autres de communautés d'agglomération, d'autres encore de communautés de communes, d'autres du département ou du centre de gestion ... De fait, cet article va dans le sens de la libre administration des collectivités territoriales : celles-ci doivent pouvoir choisir la manière dont elles souhaitent se mutualiser. La France n'est pas encore l'Union soviétique, Dieu merci

lors, compte tenu de l'importance croissante du numérique dans notre société, de son impact et des enjeux qui s'y rapportent- dématérialisation des services, inclusion numérique, ouverture, sécurisation et protection des données -, il est assez surprenant

obligation nouvelle ; c'est une incitation forte du législateur à ce que les élus locaux s'emparent eux-mêmes de cette question de la stratégie

collectivités ont d'abord besoin de s'adapter, de passer la première étape avant d'aborder la seconde. La commission ne souhaite donc pas multiplier les documents de planification obligatoires à leur charge, du moins aujourd'hui.

des plaques d'immatriculation pour produire des informations statistiques à des fins de régulation du trafic routier ou d'organisation de la mobilité. Pour l'heure, cette technologie est réservée aux forces de police et de gendarmerie, à des fins de prévention ou de répression d'infractions pénales particulièrement graves, comme le terrorisme, la criminalité organisée, contrebande en bande organisée, le vol et le recel de véhicules, ou encore d'infractions douanières. La loi de modernisation de la justice du XXIsiècle a prévu d'étendre son utilisation à la constatation des infractions au code de la route, mais on attend toujours le décret d'application. Il ne paraît pas opportun d'étendre aujourd'hui l'utilisation d'une technique aussi intrusive à des fins de gestion de la mobilité,

absolu des prérogatives du Parlement, le Gouvernement a décidé de déposer un projet de loi permettant de mettre en oeuvre le règlement européen et de transposer la directive, sans solliciter d'ordonnance pour ce faire. Les assemblées sont donc saisies des dispositions législatives nécessaires pour assurer la conformité de notre droit national à cette nouvelle réglementation européenne ; aucun des choix politiques ou juridiques pour ce faire n'est ainsi soustrait à l'appréciation du Parlement. Le Gouvernement souhaite naturellement que soit respectée l'échéance du 25 mai 2018, date à laquelle le règlement européen sera applicable. C'est pourquoi il a fait le choix d'un texte très resserré, et non d'une réécriture de l'ensemble de la loi de 1978,

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement sollicite du Parlement une habilitation pour codifier les modifications apportées à notre droit par ce projet de loi dans la loi fondatrice de 1978. Ainsi, nous offrirons un cadre juridique lisible, sécurisé et stable

que le Parlement sera amené à faire lors du vote du texte. Non seulement le Gouvernement s'y engage, mais cet engagement résulte des termes mêmes de l'habilitation qui vous est soumise. Le Conseil d'État, dans son avis sur le projet de loi, a validé cette démarche, tout en réduisant le délai d'habilitation à six mois. Vous proposez quant à vous, madame la rapporteur, de ramener ce délai à quatre mois. L'habilitation sollicitée permettra

L'ordonnance permettra également de mettre en cohérence l'ensemble de la législation applicable à la protection des données à caractère personnel, afin d'apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et omissions résultant de la présente loi et abroger les dispositions devenues sans objet. La démarche adoptée par le Gouvernement consiste donc à soumettre au Parlement les questions posées par la transcription dans notre droit des nouvelles règles européennes sans avoir à employer son temps, que l'on sait précieux, à opérer une codification qui ne pourra qu'intervenir à droit constant, compte tenu des termes mêmes de l'habilitation et de la nécessité d'offrir aux citoyens un cadre juridique clair et lisible.

et de sécurité juridique pour les acteurs économiques. À ce titre, le Gouvernement vient de s'engager devant le Sénat à offrir un cadre juridique lisible consistant en une simple codification, sans rien changer aux décisions du Parlement. Je pense évidemment à nos collectivités territoriales et à nos TPE et PME. Il s'est également engagé à informer régulièrement le Parlement de l'avancement du projet d'ordonnance. Le présent sous-amendement vise à prendre acte de ces engagements donnés au Sénat et à encadrer à double titre l'habilitation sollicitée. Sur le fond, il a pour objet de préciser expressément que l'ordonnance ne pourra modifier les équilibres auxquels sera parvenu le Parlement.

je ne m'attarderai pas, puisque j'accepte tout à fait la modification que vous proposez. Vous me permettrez d'être un peu plus réservée sur le second point de votre sous-amendement, c'est-à-dire quant à la durée dans laquelle vous souhaitez que soit inscrite la démarche de rédaction

que nous avions envisagé initialement, dix-huit mois, a déjà été ramené à six mois par le Conseil d'État. J'entends bien évidemment la nécessité dont vous faites état de procéder le plus rapidement possible

Il convient donc, tout d'abord, que le texte soit définitivement voté pour que nous puissions disposer d'une vision d'ensemble pour procéder à la remise en forme cohérente de la loi de 1978, sans remettre en cause- je le répète et, dorénavant, ce sera écrit écrit grâce à vos propositions -les choix fondamentaux réalisés dans le projet de loi, de façon à garantir une meilleure accessibilité de l'ensemble du droit. Il nous faut également procéder

Nous avions rejeté, en commission, le principe même de cette ordonnance. Le texte de la commission des lois n'en porte plus la trace.

ordonnance s'apparente à un exercice de codification, même s'il ne s'agit pas d'un code : il s'agit d'intégrer à la loi de 1978 Informatique et les libertés des dispositions éparses, en veillant à leur cohérence, et cela sans ajouter à ce qui sera le droit positif après la promulgation de la loi. Nous comprenons bien l'intérêt de cette démarche et la nécessité d'une plus grande lisibilité pour ceux qui ont à appliquer la loi. Quand nous avons défendu les collectivités territoriales qui se voient assigner de nouvelles responsabilités, nous avons naturellement pris en compte la nécessité pour elles de disposer de textes lisibles. C'est pourquoi nous sommes prêts à faire mouvement-

au Sénat l'adoption de l'amendement du Gouvernement si le sous-amendement de la commission des lois n'est pas préalablement adopté, et cela sans modification.

pas y voir un consentement à des ordonnances menaces que nous récusons de toutes nos forces.

Je le dis en tant que membre de la CNIL, mais aussi et surtout eu égard aux utilisateurs, aux usagers et aux gestionnaires de données. Je peux paraître

La commission des lois a réintroduit l'article 48 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui avait été abrogé par l'Assemblée nationale.

Cette lecture a d'ailleurs été confirmée par les lignes directrices relatives au droit à la portabilité des données qui ont été adoptées par le groupe de travail « G 29 » sur la protection des données, lesquelles adoptent une interprétation très large de la notion de portabilité des données personnelles. Les dispositions issues de l'article 48 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique doivent donc être supprimées pour des raisons de cohérence et de sécurité juridique. Les opérateurs économiques partagent l'analyse selon laquelle toutes les données visées relèvent en réalité d'un seul et même régime juridique, celui de la portabilité Ce régime est d'ailleurs plus aisé à mettre en oeuvre que celui des données non personnelles, puisqu'il permet une portabilité directement de terminal à terminal et une transmission des données directement d'un responsable de traitement à un autre, lorsque cela est techniquement possible. Pour toutes ces raisons,

? Cet amendement vise à supprimer le droit à la récupération et à la portabilité des données non personnelles introduit dans le code de la consommation par la loi pour une République numérique. Certes, la portabilité des données personnelles est désormais bien assurée dans le cadre du RGPD. C'est l'un des nouveaux C'est l'un des nouveaux droits introduits par le règlement, et il faut s'en réjouir. Reste que ce droit ne concerne que la portabilité des données personnelles. Le droit à la récupération et à la portabilité des données non personnelles est différent ; il est uniquement prévu par le code de la consommation. Il s'agit, concrètement, de faciliter le passage des consommateurs d'un opérateur de services électroniques à un autre, à savoir l'exportation de mails, de fichiers, de. Il s'agit d'un réel enjeu non seulement pour les consommateurs, mais aussi pour la concurrence.

Les consommateurs bénéficient désormais d'un droit de récupérer leurs données, puisque les fournisseurs de services de communication au public en ligne ont une obligation de mettre en place une fonctionnalité permettant au consommateur de récupérer " l'ensemble de ses données un périmètre qui inclut des données personnelles, pour lesquelles la CNIL est compétente, et des données non personnelles, pour lesquelles la DGCCRF est compétente. » Ensuite, la direction des affaires civiles et du sceau- mois de février 2017 aux députés rapporteurs de la mission d'information sur les incidences des nouvelles normes européennes en matière de protection des données personnelles sur la législation française, a elle-même confirmé que les deux régimes de portabilité étaient bien distincts et « cohérents ». À la page 87 de cet excellent rapport parlementaire, rapport parlementaire, il est précisé : « Les données n'ayant pas un caractère personnel visées par [le droit à la portabilité de la loi pour une République numérique] sont les données anonymes au sens du règlement [ ...] Ces données étant situées hors du champ d'application du règlement, les deux régimes de portabilité sont [ ...] compatibles. ...ces deux régimes semblent cohérents. »

Dans le cadre du projet de loi qui vous est soumis, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement a souhaité maintenir une formalité préalable particulière pour les traitements qui nécessitent l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, le NIR. Ce type de traitement est ainsi autorisé par un décret pris après un avis motivé et publié de la CNIL, qui définit les catégories de responsables de traitement et les finalités pour lesquelles ces traitements peuvent être mis en oeuvre. Ce décret-cadre a vocation à recenser l'ensemble des traitements existants utilisant le NIR. Dans un objectif de sécurité Dans un objectif de sécurité juridique pour les administrations de l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés, il est prévu au travers de cet amendement que les traitements qui n'auraient pas été mentionnés dans l'une des catégories de responsables de traitement et pour une des finalités définies dans le décret-cade ne deviendront pas illégaux le 25 mai 2018 de ce seul fait. J'insiste sur l'expression « de ce seul fait ». En effet, ces traitements restent soumis en tout état de cause à l'ensemble des autres obligations qui découlent de la loi et du règlement de 2016. Ainsi, les traitements qui ont été autorisés par acte réglementaire ou par la CNIL avant le 25 mai 2018 ne sont pas soumis jusqu'à leur modification, et au plus tard jusqu'au 25 mai 2020, à l'obligation d'être mentionnés dans le décret-cadre. Quel est l'avis de la commission ?

de l'effacement de droit des données inscrites au traitement d'antécédents judiciaires, dont la conservation est interdite. En effet, l'effacement des données est naturellement de droit, sans nécessiter d'autre fondement légal que la loi de 1978. Affirmer un droit à l'effacement spécifique au TAJ conduit à créer une disposition législative spéciale, alors qu'elle ne déroge en réalité pas au droit commun. Un tel ajout me semble dès lors inutile et susceptible par ailleurs de générer un, sauf à devoir modifier l'ensemble des traitements autorisés pour rappeler ce principe.

Néanmoins, les services semblent visiblement avoir tendance à ne pas vouloir participer à l'effacement de ces données. Alors que nous n'avons aucune garantie sur la future articulation entre les dispositions générales et spécifiques de la loi de 1978, il me semble nécessaire d'affirmer, de manière spécifique pour le TAJ, que l'effacement des données illégales est de droit. Je rappelle que, en application des dispositions votées à l'article 19 du projet de loi, notamment celles qui concernent l'article 70-21, cet effacement ne semble pas être consacré entièrement de plein droit. La précision apportée en commission reste donc utile. au 31 décembre 2017, que 14 396 267 personnes étaient enregistrées dans le TAJ en tant que mises en cause et 42 028 933 en tant que victimes.

du délai de réponse des magistrats compétents pour traiter des demandes de rectification ou d'effacement des données inscrites au TAJ. En effet, la plupart des parquets ne sont actuellement pas en mesure de respecter le délai d'un mois. En outre, cette extension du délai se justifie par la très probable augmentation du nombre de demandes qui résultera des possibilités nouvelles d'effacement anticipé permises par le projet de loi, en l'absence de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire.

au ministère public ou à une juridiction pour statuer sur toute demande qui lui est adressée. Il me semble dès lors à la fois cohérent et nécessaire de rétablir l'allongement d'un à deux mois du délai de réponse des magistrats compétents. Quel est l'avis de la commission ?

la garde des sceaux. et à rétablir ainsi le principe d'une mention de ces décisions au TAJ, sauf décision d'effacement du procureur. En effet, la situation des personnes ayant fait l'objet d'un classement sans suite ou d'une décision de non-lieu ne peut pas être assimilée à celle des personnes ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement. Si une telle décision définitive de relaxe ou d'acquittement interdit toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits, tel n'est pas le cas d'un classement sans suite ou d'un non-lieu. En effet, les poursuites peuvent toujours être entreprises tant que l'action publique n'est pas éteinte, notamment en cas de nouvelles charges découvertes après un non-lieu. Le classement sans suite ne résulte pas nécessairement d'une absence d'infraction ou d'une insuffisance de charges. Il peut intervenir en opportunité, alors que l'infraction a bien été commise, notamment à la suite de l'exécution d'une mesure alternative aux poursuites, comme un rappel à la loi, une orientation sanitaire, un éloignement du domicile conjugal ou une médiation pénale. Ainsi, des données liées à la commission de violences conjugales ayant donné lieu à un classement sans suite après exécution d'une médiation pénale doivent, par principe, rester inscrites au TAJ, et non pas être effacées comme le prévoit le texte dans sa version issue des travaux de la commission des lois. Ces données ne seront cependant utilisées que pour des finalités judiciaires, car elles feront alors l'objet d'une mention qui en interdit l'accès, dans le cadre d'enquêtes administratives, ce qui garantit les droits de la personne.

Il convient, en effet, de pouvoir conserver des informations concernant des non-lieux ou des classements sans suite dans la perspective d'une réutilisation à d'autres fins ultérieures. Néanmoins, le texte de la commission n'obère pas cette possibilité. Il pose seulement un principe : sauf décision contraire, le principe doit être l'effacement des données et l'exception le maintien des données.

ainsi rédigé : « L'ensemble des personnes précitées doit veiller à l'authenticité des pièces produites dans le cadre d'une demande. À cette fin, elles disposent d'un accès au répertoire national mentionné à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale et aux avis d'imposition des demandeurs. Il leur est également possible de solliciter directement auprès de leur employeur la copie de leur contrat de travail ainsi que les trois dernières fiches de paie. paie. » Cet amendement a pour objet d'utiliser une des marges de manoeuvre mentionnées au f du 1 de l'article 6 du règlement général sur la protection des données. Les collectivités territoriales et les bailleurs sociaux pourront désormais contrôler l'authenticité des pièces qui leur sont communiquées dans le cadre d'une demande de logement locatif social. Ainsi, une telle possibilité offerte au responsable de traitement répond à deux intérêts légitimes que sont la lutte contre la fraude et l'égalité de

Il autoriserait ainsi désormais l'accès des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux au Répertoire national commun de la protection sociale, qui est un traitement de données sensibles puisqu'il concerne le numéro de sécurité sociale, l'un des traitements les plus protégés, au contrat de travail des demandeurs de logements sociaux et à leurs trois dernières fiches de paie. Ces informations pourraient même être directement obtenues auprès de l'employeur. La commission n'y est pas favorable. Cet amendement ne s'articule pas bien avec les autres dispositions du texte. Le projet de loi encadre désormais bien plus strictement l'usage du numéro de sécurité sociale ; il s'agit d'une donnée sensible, très identifiante. Les données contenues dans le Répertoire portent en outre sur des informations sensibles qui concernent des publics particulièrement vulnérables. À rebours de l'intention protectrice du projet de loi, le présent amendement élargirait l'accès au Répertoire national pour de nouvelles finalités, sans prévoir de garanties spécifiques en contrepartie. En outre, cet amendement met à la charge des collectivités territoriales et des bailleurs sociaux une nouvelle obligation de vérifier l'authenticité des pièces produites par les demandeurs d'un logement locatif social. Des bailleurs sociaux nous ont fait part de leur hostilité au dispositif et de leur crainte des contentieux qu'occasionnerait pour eux cet amendement. La commission demande

C'est un outil de justice, tout simplement, que de ne pas donner un logement social à quelqu'un qui ne produirait pas des pièces authentiques. Je ne comprends pas ces pudeurs.

années, produisant des coûts très importants pour les départements, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, avec des enfants, des familles en difficulté

des parlementaires de déposer des amendements. Les raisons pour lesquelles un certain nombre d'amendements ont été refusés, dans une loi pourtant qui portait sur la confiance

à l'usage aléatoire de l'article 45 de la Constitution. Personne ne nous le demande ; le Sénat est seul responsable dans cette affaire.

qui méritait un débat. D'ailleurs, le fait que beaucoup d'entre vous se soient inscrits dans ce débat le prouve ... Je voudrais saluer les propos de M. Savary comme de Mme Primas,

telle difficulté à résoudre suppose d'inscrire la réflexion dans un cadre qui lui soit propre, d'autant plus que la question de l'insolvabilité de compatriotes en situation précaire se pose non seulement pour les bailleurs sociaux, mais aussi pour beaucoup de propriétaires, souvent eux-mêmes impécunieux, qui sont confrontés à une pratique de concitoyens en difficulté pour lesquels le loyer est la variable d'ajustement la plus facile à utiliser pour faire face au quotidien, en éloignant le versement de leur dette de logement. Aussi, la recherche des moyens pour les bailleurs sociaux, comme pour les propriétaires privés, de rétablir un équilibre qui s'est parfois rompu me paraît totalement légitime. Notre collègue Henri Leroy ne pouvait pas être présent ce soir, mais j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec lui de sa proposition, qui est inspirée par des motifs que je crois dignes d'être pris en considération. Après avoir dit cela, je suggère que nous reprenions ce débat avec la commission des affaires sociales et avec la commission des affaires économiques. Il viendra suffisamment vite pour que l'on ne regrette pas de l'avoir différé ce soir.